meilleure clarté de nos débats, je souhaiterais que soient appelés en priorité, à l'issue de nos discussions sur l'article 1 A, les articles 3

ne voulons pas supprimer l'article 1 A, car nous sommes favorables à l'établissement d'une cartographie des zones propices à l'implantation des énergies renouvelables pour l'ensemble des territoires,

cohérent, fondé sur trois principes. D'abord, l'atteinte de l'objectif zéro carbone en 2050 implique une mise en oeuvre planifiée des projets d'énergies renouvelables résultant de la PPE.

Ensuite, le volet « énergie » des Scot permet d'organiser, dans le dialogue entre la région, les EPCI et les communes, la planification territoriale nécessaire, inscrite dans les PCAET.

ne l'oublions pas -pour mener la procédure de concertation préalable auprès du public.

des Scot. La planification est une bonne chose. En matière d'urbanisme, dans notre pays, chaque commune définit la destination des zones à urbaniser. En matière d'éolien, faire du zonage

de difficultés locales qui font que les populations se divisent et que les maires s'arrachent les cheveux- quand il leur en reste. Je vous suivrai, mais j'ai besoin d'être confortée dans ce que je crois avoir compris. La parole Monsieur le rapporteur

aujourd'hui jusqu'à six fois plus d'énergie annuelle qu'une éolienne construite en 1995 et certaines cellules photovoltaïques sont deux fois plus efficaces qu'il y a dix ans. Il est donc nécessaire d'encourager le renouvellement des parcs éolien et photovoltaïque les plus anciens, afin d'améliorer leur rendement. Ce potentiel est largement sous-estimé, notamment en matière de photovoltaïque, puisque 6 000 centrales solaires de première génération sont encore en activité. Le renouvellement de la centrale solaire du centre postal de la Millière dans le XI arrondissement de Marseille est un exemple à suivre. Ce bâtiment était équipé, depuis 2009, de plus de 2 500 panneaux photovoltaïques. Après avoir remplacé ces panneaux, la production globale de la centrale a augmenté de 32 %. Le renouvellement des centrales permet également de développer une filière du réemploi et de l'occasion, puisque 75 % de ces anciens panneaux seront reconditionnés et réintroduits sur le marché. Ainsi, les objectifs régionaux du développement des énergies renouvelables doivent tenir compte du potentiel du renouvellement des parcs éoliens et solaires. Cela permettra d'augmenter la production d'énergie renouvelable, sans consommer d'espace supplémentaire.

dans ce projet de loi, dès l'article 1 A, que les mesures en faveur du développement des énergies renouvelables doivent s'articuler, dans une démarche globale et durable, avec la protection de l'environnement et la préservation de nos écosystèmes et de notre biodiversité. Quel Quel est l'avis de la commission ? 1 A. En visant le « patrimoine commun de la Nation », il est fait référence à la notion inscrite à l'article L. 110-1 du code de l'environnement : « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants

à l'instar des autres collectivités, destinataires du document élaboré par l'autorité compétente de l'État, identifiant les objectifs indicatifs de la puissance à installer sur les territoires. En effet, depuis en oeuvre du Grenelle de l'environnement, le département est un acteur à part entière de la transition énergétique des territoires. L'échelon départemental permet de nouer un dialogue de proximité et de traduire des objectifs relatifs aux EnR ancrés dans les territoires.

d'énergies renouvelables sur son territoire,

climat-air-énergie, qui est un outil de planification à la fois statistique, stratégique et opérationnel permettant d'accompagner les communes et les EPCI, mais aussi les entreprises dans la mise en oeuvre des orientations stratégiques

émet un avis défavorable,

ces deux amendements identiques sont satisfaits par les dispositions intégrées dans l'article 1 A en matière de planification. D'ailleurs, les comités régionaux de l'énergie, créés par la loi Climat et résilience, il y a un an, intègrent

Je retire l'amendement, madame

les outre-mer dans les zones qui seront identifiées par le décret en Conseil d'État. Pour ces territoires, les problématiques de dépendance énergétique et d'utilisation des ressources environnementales sont en effet fondamentales. Dans les départements et régions d'outre-mer, la production électrique dépend majoritairement du pétrole et du charbon, alors que le potentiel des énergies renouvelables est très important.

de la multiplicité des acteurs qui interviennent désormais dans ce nouveau champ d'activité. Il s'agit donc par cet amendement de veiller à ce que soient précisés par décret les moyens mis en oeuvre pour cette régulation et les possibilités de recours pour les citoyens ou les collectivités locales qui seraient impactés par les décisions prises en vertu de cet article 1 A. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l'alinéa 20. Je confirme qu'il faudra que le décret puis des instructions ciblées du Gouvernement aux services déconcentrés précisent les conditions d'application de cet article, notamment les éléments que vous mentionnez.

Ce texte est essentiel parce qu'il prévoit de réelles simplifications en matière d'urbanisme. Notre assemblée a toujours alerté sur la lourdeur des procédures, qui est l'un des principaux obstacles à l'émergence des projets. Le développement des énergies renouvelables passera, certes, par de grands projets, mais surtout par la multiplication de petits projets au coeur des territoires. Nous avons cependant prévu plusieurs garde-fous, afin de garantir que la simplification ne se traduise par exemple, que toute évolution du zonage fasse bien l'objet d'une réflexion approfondie et résulte du choix des élus. Surtout, nous avons exprimé clairement notre ligne rouge : nous ne voulons pas d'interventionnisme direct de l'État dans le coeur des documents de planification des collectivités. J'espère que le Gouvernement a entendu ce message, porté sur toutes les travées. À la marche forcée centralisatrice, nous avons préféré des outils décentralisés à la main des collectivités. C'est pourquoi nous avons renforcé le volet « énergies renouvelables » des Scot, et proposé que ceux-ci puissent délimiter les zones d'implantation prioritaire des sites d'énergies renouvelables. Nous améliorons ainsi la planification par les élus, en nous appuyant sur des outils et des modes de gouvernance déjà bien éprouvés, connus et pratiqués par les élus, et fiabilisés juridiquement. Nous avons également ajouté un avis conforme des conseils municipaux, sans créer d'obligation ni de procédure additionnelles.

par les collectivités, et mieux encadrer l'implantation des autres projets. Enfin, cet article 3 est essentiel parce qu'il prévoit les articulations nécessaires avec l'objectif « zéro artificialisation nette ». Vouloir développer les énergies renouvelables en France sans se préoccuper de la mobilisation du foncier est une hypocrisie. Notre commission a ainsi proposé plusieurs solutions

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet article tend à simplifier la procédure de modification des projets d'aménagement et de développement durable.

C'est au motif d'une célérité justifiant aussi, apparemment, l'absence de consultation de certaines instances que vous introduisez une disposition pouvant être néfaste pour l'écologie et la démocratie locale. En d'autres termes, vous voulez faire vite et plus, et donc vous bâclez. Nous n'en sommes pas surpris, car cela devient, hélas, une habitude. Je tiens cependant à rappeler que, si le Conseil constitutionnel n'a malheureusement pas consacré ce principe de non-agression du droit de l'environnement, il a néanmoins dressé un cadre dans sa décision du 10 décembre 2020. Ainsi, en tant que législateurs, nous avons le devoir de prendre part de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, conformément à l'article 2 de la Charte de l'environnement. Madame la ministre, nous savons

peuvent être identiques et aussi lourdes que celles requises pour l'installation du projet lui-même. Cet amendement vise donc à simplifier et accélérer les procédures administratives permettant de réaliser des opérations de reconnaissance préalable, destinées à vérifier la faisabilité d'un projet d'énergies renouvelables ou de stockage d'électricité, lorsque les opérations doivent être effectuées sur des espaces remarquables dans le cadre de la loi Littoral. Je précise enfin que la simplification proposée existe déjà pour d'autres secteurs d'activité. L'amendement n° 520 n'est pas soutenu. Quel est des affaires économiques ? Nous voyons trois difficultés majeures à autoriser, en bloc, les opérations de prospective et de reconnaissance au sein des espaces remarquables et des milieux protégés par la loi Littoral. D'abord, une autorisation générale, et non au cas par cas en fonction des projets, me semble insuffisamment justifiée au regard des enjeux environnementaux. Il faut prévoir une modalité de contrôle, des garde-fous. Ensuite, la réduction de la consultation du public dans des espaces qui font justement l'objet d'une protection renforcée me semble risquée du point de vue de l'acceptabilité des projets. Surtout, il me semble que les collectivités compétentes ne seraient pas forcément toujours d'accord avec ces opérations de prospection,

Cet amendement vise à introduire diverses coordinations juridiques et rédactionnelles, afin de tenir compte des modifications de l'article intervenues lors de l'examen en commission et d'harmoniser la rédaction des différentes mesures, en prenant notamment en compte l'extension du champ de l'article au stockage des énergies renouvelables.

Cet amendement vise à supprimer l'hydrogène bas carboné, et les installations qui en découlent, de la liste des énergies pouvant faire l'objet d'une procédure de modification simplifiée dans les documents d'urbanisme locaux prévue dans le présent article. Si nous souhaitons le renforcement de la filière de l'hydrogène renouvelable, fabriqué à partir de l'électricité provenant uniquement des sources d'énergies renouvelables et qui, de fait, peut être un vecteur de la transition énergétique, l'hydrogène bas-carbone est produit soit à partir d'énergies fossiles avec captation de carbone, soit à partir d'électricité provenant de l'énergie nucléaire. L'hydrogène bas carboné ne peut donc pas être considéré comme une énergie renouvelable, et n'a pas sa place dans ce projet de loi.

à revenir sur les mesures adoptées dans le cadre de la loi Climat et résilience et précisées par les deux décrets du 29 avril 2022. Ces modifications ne sont pas nécessaires, dès lors que la plupart des installations de production d'énergie renouvelable- éolienne et photovoltaïque notamment -et des ouvrages de raccordement à un réseau public de transport (RPT) d'électricité ne seront, en pratique, pas comptabilisés dans le cadre de l'objectif « zéro artificialisation nette En effet, je veux le rappeler très concrètement, avant 2031, une installation photovoltaïque au sol ne sera pas considérée comme une consommation d'espace

aux méthaniseurs, le plus souvent installés dans un espace agricole, à côté d'une unique ferme ou de quelques bâtiments agricoles, ils ne créent pas ou n'étendent pas, sauf exception, un espace urbanisé. Pour toutes ces raisons, je vous propose de soutenir cet amendement qui vise à simplifier la rédaction du projet

l'objectif « zéro artificialisation nette ». Le Gouvernement ne peut ignorer l'impact qu'aura cet objectif sur la capacité à mobiliser le foncier en faveur des EnR : il est temps de résoudre ces injonctions contradictoires. Nos articulations sont proportionnées et nécessaires, et apportent des outils aux collectivités. Elles seront d'ailleurs complétées par nos collègues de la

à l'échelle communale, intercommunale ou régionale, est comptabilisé nationalement et fait donc partie de l'enveloppe globale du ZAN. À cet égard, j'aimerais entendre Mme la ministre, car ce n'est pas du tout la même chose

Le texte prévoit désormais que les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer des objectifs et délimiter des zones d'implantation prioritaires en matière d'énergies renouvelables. C'est un point très positif de l'évolution du texte, car, chacun d'entre nous a pu le constater, la multiplication d'implantation de projets de façon désordonnée et non concertée a entraîné des incompréhensions et des rejets de la part des populations. L'absence de cadre cohérent a par ailleurs laissé les maires seuls face à des choix énergétiques qui engagent pourtant l'avenir de tout un territoire. Or le déploiement des énergies renouvelables, leur nature, leur localisation et leur impact doivent nécessairement s'inscrire dans une stratégie territoriale pensée avec les élus locaux, et s'accompagner d'une meilleure implication des habitants. Notre amendement vise à aller plus loin dans la rédaction issue des travaux de la commission. Il renforce davantage encore le volet « planification énergétique » du Scot en cohérence, bien sûr, avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, et en articulation avec les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Ainsi, le Scot fixerait obligatoirement les orientations et objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Il identifierait les zones propices à l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Le Scot mettrait ainsi mieux en perspective le potentiel de développement d'un territoire, ses contraintes locales et la prévention des conflits d'usage, particulièrement avec la production agricole et l'exploitation forestière. Il organiserait mieux l'articulation avec les autres politiques sectorielles, notamment celle du foncier. Ce pilotage renforcé à l'échelle du Scot permettrait également de mieux associer les citoyens, d'accompagner l'émergence de nouvelles solidarités territoriales et une répartition plus équilibrée des installations. L'adoption de cet amendement nous permettrait de développer un débat plus apaisé sur le sujet.

et en prévoyant des bonus dans les appels d'offres pour ces zones. Vous l'avez compris, le Gouvernement souhaite donner plus de poids à la planification locale réalisée par les intercommunalités,

de partenaires de la politique énergétique de notre pays. Nous le ferons, par exemple en fléchant des appels d'offres sur ces zones prioritaires et en faisant en sorte que, dans les appels d'offres plus larges,

permettront de lever des obstacles au développement des énergies renouvelables, en favorisant tous les élus qui s'engagent fortement dans la planification territoriale et écologique,

les collectivités qui le souhaitent peuvent, comme aujourd'hui, avoir recours aux Scot pour encourager le développement des EnR. Nous ne voulons pas transformer cette possibilité en obligation, notamment pour prendre en compte les territoires dans lesquels la gouvernance du Scot est moins performante

le gaz, avec des opérations individuelles ou semi-collectives entre plusieurs agriculteurs ou industriels.

important, car les conseillers municipaux sont représentatifs de l'ensemble de la population : ils portent la parole de celles et de ceux qui sont favorables

et j'en suis arrivé à la conclusion que le maire peut, avec son conseil municipal, s'opposer

Un point me paraît important : on parle de l'implantation des énergies renouvelables et de la planification, mais on ne fait pas de l'éolien ou de la géothermie n'importe où sur le territoire ... Il faut des études

j'aimerais vraiment qu'une réponse soit donnée à la question de notre collègue du groupe CRCE : le dispositif qui est en train d'être élaboré ici, sur proposition de la commission, permet-il, oui ou non, d'accueillir

la commune sera appelée à donner son avis, et éventuellement à refuser le zonage. La question est la suivante : si l'autorité qui a compétence pour le Scot

au règlement du PLU de « délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. » Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables, mais la transition écologique ne peut se faire sans l'engagement des communes et des intercommunalités, ce qui suppose que celles-ci soient plus impliquées dans la définition de l'avenir énergétique de leur territoire, en particulier pour le choix des énergies renouvelables qu'il conviendrait d'y développer ainsi que de leur emplacement.

peut être soumise à conditions. Cela concerne également les ouvrages de réseau public de transport et de distribution d'électricité.

qui permet d'afficher le projet de territoire de la collectivité et de définir les orientations des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que de définir les orientations générales concernant l'énergie. Les orientations d'aménagement et de programmation sont également opposables aux porteurs de projets dans un rapport de compatibilité et permettent de décliner les orientations du PADD. Le règlement du PLU peut enfin préciser finement l'insertion des projets en délimitant des secteurs dans lesquels l'implantation d'EnR d'EnR sera, pour des raisons de protection paysagère ou patrimoniale, fortement encadrée et limitée et, à l'inverse, des secteurs où ces EnR peuvent être installées de manière préférentielle. Nous disposons déjà de beaucoup d'outils

une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme permet de contourner la réalisation d'une enquête publique. La consultation se résume alors à une mise à disposition, organisée par la commune. Les zones boisées et les zones agricoles ou naturelles sont des espaces sensibles, qui contribuent au paysage, au patrimoine et à l'économie d'un territoire. Il serait impensable de transformer ces espaces sans consulter celles et ceux qui y vivent.

nette ». Les espaces forestiers permettent de produire des matériaux et des énergies renouvelables. Il est donc indispensable et essentiel de les préserver. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à supprimer les dispositions facilitant le déboisement de nos forêts. Les trois amendements

Il est nécessaire d'empêcher toute modification simplifiée du plan local d'urbanisme concernant les règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières. Ces dernières doivent faire l'objet d'une protection particulière contre l'artificialisation, ce qui suppose qu'elles ne puissent

décrit les cas de révision du plan local d'urbanisme. Le PLU doit notamment être révisé lorsque l'EPCI ou la commune décide de changer les orientations définies par le PADD ou de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. Or les projets d'installations de production d'énergies renouvelables sont précisément de nature à réduire un espace boisé

par l'illectronisme, nous ne sommes pas favorables à ce que l'enquête publique puisse être court-circuitée- lorsqu'il s'agit de zones agricoles, naturelles ou forestières. Nous souhaitons préserver la procédure standard de modification du PLU pour ces zones, qui doivent être particulièrement protégées contre l'artificialisation. Nous ne sommes pas favorables à un déclassement vers d'autres zonages plus faciles à artificialiser.

Il s'agit simplement de modifier le règlement d'urbanisme pour préciser les types d'installation autorisés et leurs caractéristiques, dans les limites fixées par la loi. De plus, De plus, la modification simplifiée assure également la participation du public et des personnes publiques associées. Nous devons faire confiance aux élus locaux pour soutenir les projets qu'ils estiment pertinents pour leur territoire et, à l'inverse, pour encadrer ceux qu'ils jugent mal conçus.

Madame la ministre,

mieux prendre en compte les enjeux de préservation du foncier agricole, les auteurs de cet amendement proposent d'instaurer une consultation pour avis simple de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans

avant que ces zones ne soient délimitées dans le Scot et n'entrent en vigueur, il faut donner aux communes et aux EPCI les moyens de réglementer les projets qui pourraient naître sur leur la loi 3DS permet de délimiter certains secteurs au sein des PLU dans lesquels les éoliennes seront soumises à condition. Nous avons voté l'extension de cette réglementation 3DS à tous les types d'EnR. Mon amendement vise donc à permettre de modifier plus rapidement les PLU pour y dessiner ces secteurs de réglementation en l'attente de l'entrée en vigueur des nouveaux Scot à la planification renforcée. Quel est l'avis de la commission

même s'il n'a aucun lien avec une installation de production d'électricité renouvelable. C'est la raison pour laquelle nous proposons de restreindre explicitement cette possibilité aux seuls ouvrages dont la construction est nécessaire pour le raccordement au réseau d'une ou de plusieurs installations de production d'électricité renouvelable, toujours dans un souci de cohérence avec l'intitulé de ce projet de loi. Quel est l'avis de la commission

Il serait donc périlleux, juridiquement comme dans la pratique, de séparer les ouvrages strictement nécessaires à tel ou tel site de production du reste du réseau, qui est une infrastructure globale.

par modification simplifiée, au même titre que les orientations du PADD, lorsque cette modification vise spécifiquement à autoriser l'implantation d'un projet de production d'énergies renouvelables. Cet article vise également à permettre la mutualisation de droit des effets des projets majeurs d'énergies renouvelables soutenus par les collectivités et par l'État collectivités et par l'État en termes d'artificialisation. Afin de border ces dérogations et d'apporter des garde-fous utiles pour la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, nous proposons que la CDPENAF puisse émettre un avis simple sur tout projet entrant dans le champ des dérogations à l'objectif zéro artificialisation nette pour les projets de production d'énergies renouvelables mis en place par le présent article. Quel économiques ? La CDPENAF est déjà automatiquement saisie lorsque la modification d'un Scot a pour effet de réduire des surfaces agricoles, naturelles ou forestières- elle peut même s'autosaisir. Je ne souhaite pas modifier dans ce texte la gouvernance plus large du ZAN, sujet sur lequel travaille actuellement la mission conjointe de contrôle créée par quatre commissions.

prévoit qu'une installation de production d'énergie photovoltaïque implantée sur un espace naturel et agricole « n'est pas comptabilisée dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée Les espaces forestiers seraient exclus de cette dérogation. Cette lecture est confirmée par le projet de décret du Conseil d'État définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre de l'alinéa précité. Ce projet de décret a été soumis à consultation en mai 2022 et n'est pas publié à ce jour. Sa notice le précise, « au sens de la loi, les installations implantées sur un espace forestier ne bénéficient pas de cette dérogation et sont donc comptabilisées dans la consommation d'espaces NAF, naturels, agricoles et forestiers ». La différence de traitement entre une installation de production d'énergie photovoltaïque sur des parcelles agricoles et une installation sur des parcelles forestières ne se justifie pas. Par ailleurs, cette dérogation pour les seuls espaces forestiers peut entraîner une mutation artificielle des parcelles forestières vers des parcelles agricoles et appauvrir les massifs forestiers.

Ce que vise la dérogation citée par les auteurs, qui a été introduite par la loi Climat et résilience, est le photovoltaïque vertueux, voire réversible, qui permet de préserver les sols et l'activité environnante. en particulier l'agrivoltaïsme, auquel nous avons d'ailleurs apporté en commission un meilleur encadrement. Or, l'installation de panneaux photovoltaïques en zone forestière engendre un tout autre impact que l'agrivoltaïsme. Défricher un espace forestier pour y installer un projet d'EnR peut être, dans certains cas, nécessaire, si la collectivité soutient ce projet. Mais il me semble alors indispensable de considérer ces aménagements comme de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces, sous peine d'encourager le défrichement. Je crains donc que les auteurs de l'amendement, en souhaitant éviter la transformation d'espaces

Il porte une proposition partagée sur de nombreuses travées, directement issue des auditions et des travaux que nous menons depuis plus d'un mois. Les associations de maires, les représentants des régions, des métropoles et des intercommunalités nous l'ont tous dit clairement : pris séparément, l'impact foncier des grands projets d'intérêt national ou européen est aujourd'hui tel que ces derniers consomment à eux seuls une grande partie des « enveloppes » attribuées aux collectivités au titre du ZAN. Dans plusieurs régions, si l'on décompte par exemple les grandes infrastructures énergétiques ou les de batteries électriques, c'est non pas de 80 %, voire davantage ! C'est intenable, d'autant que c'est souvent l'État qui est à l'origine de ces grands projets et que les collectivités n'ont pas de prise sur eux. Et pourtant, nous sommes tous d'accord, ces grands projets sont absolument essentiels

Aucun d'entre nous n'est prêt à sacrifier ces grands projets. Pour résoudre ce dilemme, qui mènera les collectivités dans l'impasse, notre amendement vise, en se limitant au champ des projets d'énergies renouvelables, comme le périmètre du texte nous y contraint, à « sortir » ces grands projets des enveloppes régionales, intercommunales et communales du ZAN. Ils seraient alors comptabilisés à part, au sein d'une enveloppe nationale. Il nous faudra, dans un second temps, poursuivre la réflexion sur le traitement de cette enveloppe nationale. Mais ce traitement séparé est absolument nécessaire, car il permettra non seulement à ces grands projets de se concrétiser, mais aussi de donner aux régions et au bloc communal suffisamment de marges de manoeuvre pour conduire, à leur échelle, le déploiement des Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ? Je remercie mes collègues membres de la commission conjointe de contrôle évoquée précédemment d'avoir présenté cet amendement, qui soulève un aspect essentiel de l'articulation entre développement des EnR et « zéro artificialisation nette Nous savons, grâce aux premiers retours des conférences des Scot, mises en oeuvre par la loi Climat et résilience, et des régions, que les objectifs ZAN seront déjà, dans certains endroits, quasiment impossibles à atteindre, si l'on ne décompte pas séparément les projets d'ampleur européenne ou nationale, qui consomment déjà la quasi-totalité des enveloppes régionales. plus grands projets, dont l'intérêt national, voire européen, est avéré, il est tout à fait pertinent de prévoir une enveloppe nationale séparée plutôt qu'une enveloppe régionale. Cela laissera aux collectivités la possibilité de mettre en oeuvre, dans leur enveloppe propre, leurs projets d'ampleur plus limitée. C'est ce que l'amendement propose, en se limitant aux grands projets liés aux EnR. Cet appel est légitime et pertinent. Je crois d'ailleurs que le Gouvernement avait donné des gages en ce sens aux régions françaises, à la suite de leurs alertes. J'y suis tout à fait favorable. C'est un premier pas vers une réflexion plus globale sur le ZAN. l'avis du Gouvernement ? cette question du zonage et du principe de « zéro artificialisation nette ». Vous le savez, une consultation des préfets de région est en cours, pour recenser les grands projets d'envergure nationale et apprécier leur potentiel impact impact sur la trajectoire de réduction de la consommation d'espace et de l'artificialisation des sols. Ces projets ne se limitent pas aux installations de production, de transport et de stockage d'énergies renouvelables. L'objet de cet amendement fait

cranter cette approche dans ce texte, qui ne concerne que les énergies renouvelables. Il est important d'avoir une approche globale sur l'ensemble de ces projets d'envergure nationale, en lien avec la mission qui travaille sur le sujet au sein du Sénat. La parole

du 22 août 2021, dite Climat et résilience. Notons qu'il est important d'avoir un dialogue constructif entre les élus et les porteurs de projets,

Ce droit de veto serait également accordé aux communes limitrophes impactées en termes de visibilité, dans le cadre de l'implantation des éoliennes terrestres. Cet article ne constitue donc en rien une mesure d'accélération de la production d'énergies renouvelables. Bien au contraire, il interdit aux porteurs de projets de déposer une demande d'autorisation environnementale ou de permis de construire en cas d'avis défavorable, alors que le conseil municipal aura statué sur le fondement d'un résumé non technique de l'étude d'impact. Il envoie un très mauvais signal aux porteurs de projets, d'ores et déjà embourbés par le manque de planification territoriale, les longs délais d'instruction et le risque de contentieux à chaque étape de la procédure. En outre, cette mesure peut engendrer des conflits entre les communes qui sont prêtes à accueillir le projet et les communes limitrophes. Elle conforte la logique « pas dans mon jardin », qui favorise le rejet des énergies renouvelables et retarde notre pays dans l'atteinte de ses objectifs en matière de politique énergétique et climatique. Nous n'avons pas besoin de cela ! Les prix de l'énergie ont déjà augmenté, leur relative stabilité en France n'est que le résultat du bouclier énergétique mis en place par le Gouvernement. Il nous faut produire plus d'énergie au plus vite, pour garantir notre sécurité d'approvisionnement, dans un premier temps, et décarboner notre mix énergétique, encore constitué à 60 % d'énergies fossiles, dans un second temps. Pour résumer, cet article tend à complexifier et à allonger la procédure d'instruction de ces projets, à rebours des objectifs du projet de loi. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

l'amendement n° 523 rectifié. Dans la foulée des deux intervenants précédents, je rappelle que le dispositif que nous avons adopté permet d'identifier des zones prioritaires, qui sont validées et approuvées par les communes. N'oublions pas que la loi Climat et résilience impose aux porteurs de projets une information préalable des maires

Il n'apparaît donc pas opportun d'instaurer un droit de veto supplémentaire, qui risque d'être juridiquement fragile. En effet, la délibération doit être motivée, et je ne vois pas sur quelle base

de la discussion, la nécessité d'inclure les maires et les citoyens dans la planification en amont et dans le développement des sites de production d'énergies renouvelables. Nous continuerons d'ailleurs de le faire et d'y veiller attentivement dans la suite de nos échanges. Cela étant dit, le dispositif adopté à l'article 3 tend à améliorer nettement la souveraineté des communes en matière d'implantation de ces sites de production d'énergies renouvelables. Il est de nature, disons-le, à nous donner satisfaction et à nous rassurer sur un sujet très sensible dans nos territoires, à savoir le pouvoir des maires.

les conseils municipaux, qu'il s'agisse de la loi Asap ou de la loi Climat et résilience, qui prévoit à la fois une information préalable et un dialogue constructif entre le porteur de projet et le conseil municipal. On nous demande maintenant de supprimer ce dispositif, au motif que le conseil municipal sera consulté par l'organisme portant le Scot lors de la définition des zones prioritaires d'implantation, qui ne sont pas des zones exclusives d'implantation, ce qui veut donc dire qu'un projet peut tout à fait être implanté dans une zone non prioritaire.

où l'on peut implanter un projet en zone non prioritaire, rien ne s'opposera à ce que des éoliennes soient implantées sur le territoire de la commune. Finalement, le conseil municipal n'aura pas pu faire valoir son avis. On nous dit également que la loi 3DS protège les conseils municipaux, puisqu'ils ont la possibilité de réglementer l'implantation d'éoliennes dans le PLU. Sauf que l'État pousse à ce que les PLU deviennent des PLU intercommunaux. Ce seront donc les conseils communautaires qui pourront se prononcer.

il importe de rechercher l'acceptation de l'éolien terrestre par les habitants concernés. L'oppression dont ils sont victimes- dominance visuelle, ombres portées, bruit, infrasons, champs magnétiques, dépréciation immobilière, etc. -suscite une opposition croissante. Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010, même si une ordonnance du 26 janvier 2017 a donné aux préfets le pouvoir d'aller au-delà. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d'actualiser les 500 mètres par-delà les approches locales devant exister dans un cadre déterminé, comme nous venons d'en débattre et d'en décider. Les nuisances éoliennes sont, dans une large mesure, fonction de la hauteur des engins, elle-même assez largement corrélée à leur puissance. En Bavière, en Pologne, la distance minimale a été fixée, depuis plusieurs années, à dix fois cette hauteur, pales comprises.

pour les petits mâts, permettra de l'allonger pour les éoliennes de deuxième génération.

pour la porter de 500 mètres à dix fois la hauteur de l'éolienne. Il vise à prévoir que cette distance soit doublée en cas de visibilité des habitations. Le développement des éoliennes a ses vertus pour la production d'une énergie renouvelable et la transition énergétique. Toutefois, elle crée aussi pour les riverains qui nécessitent une adaptation de la législation afin de réagir aux problèmes concrets posés par le développement croissant des parcs éoliens. La distance d'éloignement de 500 mètres des zones d'habitation n'est donc plus suffisante.

les infrastructures atteignent 180 mètres et grandiront très bientôt jusqu'à 220 mètres, voire jusqu'à 245 mètres, soit plus que la tour Montparnasse et bientôt autant que la tour Eiffel Par ailleurs, le risque de chute de pales ou de rupture de mât existe. Plusieurs études scientifiques ont démontré que la bonne distance entre une installation et les premières habitations devait être au minimum de dix fois la hauteur de la structure en bout de pale en cas de chute simple et de douze fois en cas de chute avec rebond.

voté la planification et la définition de zones propices au développement des énergies renouvelables. Il appartiendra aux élus locaux de définir, dans ce contexte et dans ce cadre, les distances qu'ils souhaitent voir respectées pour l'implantation d'éventuels parcs éoliens.

tous les contentieux sur les projets éoliens portent sur quatre points essentiels : les nuisances en termes de bruit, les nuisances en termes de champs magnétiques et de santé-

l'année dernière, un tiers des appels d'offres y ont été infructueux. Il ne faudrait pas que la France soit la variable d'ajustement des constructeurs d'éoliennes dans l'Union européenne. J'en viens à mon amendement. Les parcs nationaux et régionaux, qui figurent parmi les symboles de l'identité française, ont été créés avant tout pour protéger nos paysages, dont dépendent non seulement le maintien du potentiel touristique de notre pays, mais également le respect de la biodiversité. Des éoliennes ont été acceptées dans certains parcs que, pourtant, elles altèrent. Il importe de prévenir la répétition de ces erreurs. La protection doit en outre s'étendre aux communes limitrophes, car un parc entouré de hautes silhouettes l'on verrait de loin- que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du parc -ne serait plus un parc naturel national ou régional. La protection de la biodiversité nécessite également une protection effective des sites Natura 2000, réservoirs de biodiversité pour les générations futures. C'est pourquoi cet amendement vise

de ces parcs éoliens, préférant un contrôle élargi des ABF qui, je le rappelle, n'émettent un avis défavorable que sur environ 10 % des projets qu'ils instruisent. Compte tenu des propos tenus par la Première ministre devant le Sénat voilà deux ans,

autour de ceux-ci.

Le patrimoine n'est pas responsable du réchauffement climatique, je tiens à vous le dire. Aujourd'hui il faut bien comprendre qu'aucune éolienne n'est construite dans des secteurs protégés au titre des

dans les cas très précis où existe un risque de covisibilité entre une éolienne et un monument historique, l'architecte des Bâtiments de France puisse émettre

accrues et les riverains s'en plaignent. des nuisances sonores provoquées par les implantations d'éoliennes à proximité des habitations. Cette problématique essentielle est mal appréhendée par le protocole mis en oeuvre par le ministère. Avec la pollution visuelle, il s'agit pourtant de l'une des clés de l'acceptabilité. Les normes actuellement en vigueur reposent sur la notion de médiane de bruit, sans tenir compte des pics, qui peuvent largement excéder les seuils autorisés à chaque passage de pale devant le mât. Imaginez le stress que ces bruits intermittents permanents peuvent induire sur les populations environnantes. La montée en puissance des machines donne lieu à un véritable problème de santé publique et suscite un contentieux croissant que nous ne pouvons ignorer, car nous sommes responsables de la préservation de la santé de nos concitoyens.

est déjà réglementé par l'arrêté ministériel qui définit des prescriptions générales applicables aux éoliennes soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'environnement, notamment les valeurs maximales du supplément de bruit que les éoliennes sont autorisées à produire par rapport au bruit ambiant. L'étude d'impact déposée en vue de l'autorisation du parc éolien comprend une enquête acoustique indiquant de façon théorique comment ces valeurs maximales seront respectées. Le cas échéant, elle peut prévoir un bridage. Afin d'assurer la vérification concrète de ce respect, l'arrêté ministériel qui encadre les éoliennes a été modifié au mois de décembre 2021 pour imposer au 1 janvier 2022 un contrôle acoustique systématique dans les douze mois suivant la mise en service des parcs éoliens. Si le contrôle réalisé met en évidence des dépassements du supplément de bruit autorisé, des mesures de bridage sont alors ordonnées par le préfet.

Cet amendement vise à offrir au public un moyen de suivre l'avancée administrative des différents projets et de créer des indicateurs à cette fin, pour déterminer en temps réel si les simplifications que nous adoptons dans ce projet de loi sont efficaces. Quel est l'avis de la commission ?

Monsieur Montaugé,

Cet article permet la participation de sociétés d'économie mixte locales (SEML) aux communautés d'énergie renouvelable. S'il est vrai que, dans les projets d'énergie renouvelable classiques, l'actionnaire majoritaire est souvent une entreprise privée extérieure au territoire, voire située hors de France, et que la participation de collectivités territoriales ou de SEML permet un semblant de maîtrise publique, il n'en demeure pas moins qu'en élargissant un peu plus les entités participant à la production et à la fourniture d'énergie une telle disposition contribue à libéraliser le secteur de l'énergie et à nous éloigner d'un service public indispensable au bon fonctionnement des installations et, partant, à une juste distribution pour tous les usagers. Cela illustre une volonté délibérée de démantèlement d'un modèle centralisé qui a démontré son efficacité et de retour au début du siècle dernier qui, sous couvert de transition énergétique, sans nul doute à la remise en cause de l'égalité d'accès à l'énergie sur l'ensemble de notre territoire, de l'égalité de traitement des usagers ainsi que des tarifs réglementés. Pour nous, c'est une véritable remise en cause du contrat social énergétique. La transition énergétique doit être une priorité. C'est pourquoi l'État doit y consacrer les moyens nécessaires et cesser de se défausser sur l'initiative privée ou les collectivités territoriales,

Les SEML ne figurant pas parmi les membres potentiels d'une communauté d'énergie renouvelable, elles peuvent se voir refuser la participation à de telles communautés. L'article 1 D lève cette ambiguïté en permettant explicitement la participation des SEML aux communautés d'énergie renouvelable. Cette précision semble conforme aux dispositions de la directive RED

1. Le développement de l'énergie de récupération présente en effet de nombreux avantages : il permet de lutter contre le gaspillage énergétique, de valoriser une énergie qui, si elle n'était pas captée, aurait été perdue, il évite d'avoir recours à des énergies fossiles. n'émettent pas de rejets polluants supplémentaires dans notre atmosphère et elles sont économiques. De fait, lorsque le site de récupération des énergies n'est pas éloigné des bâtiments à chauffer, les coûts de production se trouvent considérablement réduits. Cette solution a le mérite de proposer une alternative crédible au renouvelable, lorsqu'elle est plus pertinente que ce dernier en valorisant nos déchets. Compte tenu de la recherche de tels projets permettraient de concilier le développement de la production d'énergies renouvelables et celui de la récupération, apportant ainsi une réponse adaptée à un besoin spécifique en fonction des ressources

En contournant l'enquête publique malgré des raisons environnementales, en confiant la détermination des modalités d'application au Conseil d'État, en pressant le rapport du commissaire enquêteur sans accorder de moyens supplémentaires aux administrations, tout cela dans des délais difficilement tenables et pour l'ensemble des énergies intégrées à ce texte, y compris les énergies pseudo-renouvelables, cet article est en complet décalage avec les attentes des associations environnementales et des citoyens en matière de respect de la biodiversité et des garde-fous existants. C'est la raison pour laquelle nous proposons de le supprimer.

qui a pour but d'accélérer le déploiement des EnR est donc très limité. Il prive de plus la population de la possibilité de participer à l'enquête publique dans de bonnes conditions, quand cela est nécessaire.

dans la conduite des enquêtes publiques et négliger l'apport que constituent leurs conclusions. La concertation, quand elle bien menée et qu'elle associe les populations en amont, n'est pas un frein au développement des EnR. Au contraire, au-delà de l'acceptabilité que vous souhaitez atteindre, les populations s'approprient les projets, limitant tout risque de recours. C'est un leurre que de s'en prendre aux enquêtes publiques pour les remplacer par un formulaire en ligne. Par ailleurs, le commissaire enquêteur joue un rôle prépondérant dans la démocratie environnementale que nous appelons

En trente jours, le commissaire enquêteur a la possibilité de retourner sur le terrain pour étudier des points de vigilance soulevés pendant l'enquête, pour interroger toute personne lui permettant de se faire un avis sur les observations recueillies, pour étudier des propositions et les observations, enfin, pour dialoguer

pour les projets visés à l'alinéa 1, qu'il pourra être passé outre l'enquête publique, même lorsque l'autorité qui organise la consultation estime que les impacts sur l'environnement, sur l'aménagement du territoire et les enjeux socio-économiques qui s'y attachent nécessitent

n° 544. Si nous sommes favorables à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, nous souhaitons que cette accélération ne se fasse pas au détriment de la participation du public. public. L'article L. 181-10 du code de l'environnement prévoit que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, la consultation du public doit être réalisée sous la forme d'une enquête publique si, en fonction de ses impacts sur l'environnement ainsi que des enjeux socio-économiques,

nous ne sommes pas certains qu'elle permettra une véritable accélération des projets, d'autre part, parce qu'elle pourrait se traduire par une moindre concertation dans les territoires et une moindre implication d'une partie de la population peu aguerrie aux nouvelles technologies de communication. Nous pensons qu'il est nécessaire de maintenir une concertation équitable de tous les publics. Lors de la phase d'enquête publique, des permanences sont organisées par le commissaire enquêteur, qui joue un rôle de médiateur pour expliquer le dossier et permettre au public de poser des questions sur le projet. Force est de constater que 17 % de la population est touchée par l'illectronisme. En supprimant la possibilité donnée aux préfets d'engager une enquête publique lorsque les enjeux environnementaux ou socio-économiques sont importants, nous risquons d'exclure une grande partie de nos concitoyens. Comme le souligne le Conseil économique, social et environnemental dans un avis récent, l'enquête publique vise « à informer le public du processus d'évaluation environnementale conduit en amont et de la concertation associée, et à recueillir ses commentaires. C'est une étape bien identifiée dans les territoires qu'il convient de maintenir, en rappelant son rôle d'évaluation de la bonne prise en compte par le porteur de projet des demandes exprimées dans la phase de concertation amont Raison de plus pour maintenir l'enquête publique lorsque des risques socio-économiques ou en matière d'environnement sont avérés. Tel est le sens de cet amendement. La